le rapporteur a largement réécrit cet article relatif à l’affichage de l’origine des produits, qui pose le principe de la mise au point d’une proposition d’affichage obligatoire que la France devra défendre devant le Conseil de l’Union européenne. Nous proposons au travers de cet amendement une version un peu plus ambitieuse,

Les consommateurs doivent avoir accès à une information transparente sur l’origine des produits qu’ils consomment. Une enquête de l’association UFC Que Choisir, publiée il y a un an, montre que l’opacité sur l’origine concerne plus des deux tiers des ingrédients dans les produits transformés qu’elle a examinés. Alors que certaines marques donnent l’origine de plus de huit ingrédients sur dix pour les plats préparés, d’autres se contentent d’informations génériques et floues du type « origine Union européenne » ou « origine non Union européenne », ou bien ne donnent aucune mention. La transparence ou, à l’inverse, l’opacité sur les étiquetages est donc bien liée à un choix de l’entreprise, et non à des raisons techniques relevant du conditionnement des produits. Par ailleurs, cette opacité a des conséquences directes sur notre souveraineté alimentaire.

à renforcer la transparence de l’origine des denrées alimentaires que les Français consomment, en précisant que leur affichage, en plus d’être obligatoire, doit être clair et lisible. L’amendement n° 886, présenté par MM. Duplomb et Menonville, au nom de la commission

Les consommateurs doivent savoir quelle part du prix de leurs achats revient réellement au producteur. L’affichage obligatoire en grande distribution, que nous proposons, leur permettra d’opérer des choix éclairés et responsables, sans différence de traitement entre producteurs européens. Les agriculteurs demandent non pas la charité, mais une juste rémunération. En rendant visible ce partage de la valeur, nous renforcerions le lien entre producteur et consommateur et encouragerions des pratiques plus équitables. Voter cet amendement, c’est défendre une agriculture durable et responsable, ainsi que ceux qui la font vivre. Ne manquons pas cette occasion de donner à la justice agricole une dimension européenne.

La filière viticole traverse une crise durable et structurelle : aléas et crises climatiques, crise de nos exportations, crise de la promotion de nos vins à l’international et crise économique en raison d’une baisse de la consommation des vins rouges. Le président des États Unis pourrait porter les droits de douane sur l’ensemble des importations à un taux de 10 % à 20 % selon les produits, ce qui est également un mauvais signal pour nos vins et nos grands crus.

de protéger et de préserver. Il me paraît donc essentiel que les consommateurs puissent identifier clairement l’origine du foie gras qu’ils achètent. Eux aussi sont attachés à la sauvegarde d’un modèle agricole vertueux pour nos territoires. Notre amendement vise donc à rendre obligatoire cette mention d’origine. Ce gage de transparence est aussi un moyen de défendre nos filières agricoles, dans le cadre d’une concurrence souvent déloyale, et de protéger nos territoires. Dans une

rapport du Gouvernement au Parlement sur sa stratégie de lutte contre l’importation illégale de produits viticoles destinés à la vente. Il s’agit ainsi de mobiliser les services de l’État, particulièrement les douanes,

de la situation permettra également d’établir une stratégie efficace pour le secteur.

sur des leviers agronomiques et sur l’optimisation des synergies naturelles. C’est pourquoi la refonte de notre système agricole ne pourra se passer d’un engagement déterminé dans le secteur de la recherche.

la mise en culture de végétaux à vocation pollinifère et nectarifère, en vue d’augmenter le volume de ressources pour les pollinisateurs et l’ensemble de la biodiversité.

en matière de budget ne peuvent affecter ce point névralgique, au risque de compromettre directement notre futur alimentaire. L’ensemble de nos productions sont concernées et attendent une solution de la part du secteur de

un rapport circonstancié permettant d’assurer un suivi par mode de production et par filière des objectifs fixés par le Parsada.

réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour attirer les futurs jeunes vétérinaires vers la médecine des champs, plutôt que la médecine des villes,…

les exploitants agricoles ont recours aux travailleurs saisonniers, qui font partie intégrante du modèle agricole. Le travail saisonnier est au cœur de la réflexion à mener pour assurer le renouvellement des générations ; il est regrettable qu’il ne soit jamais mentionné dans ce projet de loi. Afin de fidéliser cette main d’œuvre dans un secteur identifié comme étant en tension, les travailleurs saisonniers devraient être davantage incités à suivre des formations, d’autant qu’ils peuvent devenir de potentiels repreneurs d’exploitation. En outre, dans les lycées agricoles et dans les entreprises de formation, les filles ne représentent que 32 % des élèves. L’orientation des femmes vers des études générales supérieures se fait souvent au détriment du passage par une formation agricole, qui conditionne l’obtention des dotations jeunes agriculteurs ouvrant droit aux prêts bonifiés et aux autres subventions. La complexité des trajectoires d’installation des femmes, à la différence des processus d’installation des hommes, est aussi fortement génératrice d’exclusion. Finalement, l’accès précoce des femmes à la profession demeure rare et répond souvent à des impératifs familiaux,

Le présent amendement vise donc à donner de la visibilité à ces travailleurs en les intégrant dans les dispositifs de formation. Quel

de l’article 2, relatif à l’atteinte des objectifs de nos politiques d’orientation et de formation agricoles. Depuis 2014 et le lancement d’un premier plan Enseigner à produire autrement, l’enseignement agricole tente de s’approprier les principes de l’agroécologie. En 2020, ce plan a été élargi et s’intitule désormais Enseigner à produire autrement pour les transitions et l’agroécologie. Le succès de cette démarche est aujourd’hui reconnu et de nombreuses initiatives d’innovation pédagogique et de formation des enseignants ont été engagées. Le présent amendement vise à reconnaître le succès de ce plan en

explicitement référence. En commission, les rapporteurs ont rejeté cette proposition, estimant qu’il n’apparaissait pas pertinent de se référer uniquement à ce plan. Or nous précisons bien qu’il s’agit « notamment », et non « exclusivement », de s’y référer.

le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire à l’horizon 2030. Il précise que les compétences visées doivent porter sur l’entrepreneuriat, la gestion d’entreprises, le management, le numérique et les techniques agronomiques. Dès lors que l’on choisit de lister ainsi certains domaines de compétences, nous estimons

des nouveaux actifs de l’agriculture et de l’agroalimentaire en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique. Je rappelle que 30 % à 50 % des candidats à l’installation agricole souhaitent le faire en agriculture biologique. Vous le savez, celle ci repose sur un savoir agronomique nettement plus poussé et sa pratique exige des compétences

Les derniers brevets de technicien supérieur agricole rénovés seront ainsi mis en œuvre à la rentrée 2025. Ces rénovations prévoient un développement des compétences en matière de transition agroécologique et climatique, lesquelles seront particulièrement précieuses pour tous les apprenants lors de leur insertion dans le monde du travail.

transformation et commercialisation de l’enseignement agricole public, et sont inégalement réparties selon les territoires et les cursus. Il est donc nécessaire de conforter cet enseignement. Les formations agricoles manquent en effet d’une approche technique de l’agroécologie permettant véritablement

cet amendement, notre collègue Michel Masset souhaite réintroduire, dans nos objectifs programmatiques en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation, la montée en compétences en matière de transition agroécologique, aux côtés des compétences mentionnées dans l’alinéa visé.

rectifié et vise à inscrire dans la loi que l’augmentation du niveau de diplôme en agriculture doit passer par un renforcement des compétences en matière de transition agroécologique de nos modes de production. Comme nous l’avons déjà rappelé à plusieurs reprises, nous militons en faveur d’un virage agroécologique de notre modèle agricole, qui devra nécessairement passer par l’acquisition de nouvelles compétences en lien avec les effets du changement climatique. Pour ce faire, nous devons encourager une offre de diplômes rénovée et adaptée, qui prenne davantage en compte ces enjeux. Il serait impensable d’enseigner l’agriculture aujourd’hui comme nous le faisions dans les années 1980. Nous savons que les rapporteurs n’apprécient pas le terme « agroécologie

S’adapter à une situation n’est pas exactement superposable au mot « transition ». S’adapter, c’est subir une situation et s’y

car ils vont utiliser moins d’intrants et moins d’eau, ils vont sélectionner des plantes adaptées au changement climatique et véritablement opérer une mutation de leurs pratiques culturales à la nouvelle donne climatique qui s’impose à eux. L’adaptation, quant à elle, suggère quelque chose de plus passif

pour les orienter vers les solutions qui concourent réellement à la souveraineté alimentaire et à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. La vision des rapporteurs et, hélas ! du Gouvernement d’une agriculture fondée sur l’innovation technologique et l’investissement privé, au détriment de l’emploi agricole, de l’autonomie des agriculteurs et de la biodiversité, favorise très clairement les grandes exploitations. Si l’on prend en considération les connaissances scientifiques actuelles en matière agronomique, climatique et écologique, il apparaît au contraire que les pratiques agroécologiques seront les moins coûteuses et les plus efficaces face au changement climatique, ainsi que pour améliorer les conditions de travail

à l’alinéa 11 de l’article 2, relatif aux domaines dans lesquels il est nécessaire d’amplifier nos efforts en matière de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances, que l’identification de nouvelles solutions techniques et scientifiques doit porter

pourtant présent dans le texte de l’Assemblée nationale à ce même alinéa. Nous saurons être têtus et proposerons de réintroduire partout où il le faudra la notion de transition agroécologique, qui nous semble essentielle,

d’amplifier nos efforts en matière de recherche, d’innovation et de diffusion de connaissances : ceux ci doivent porter notamment sur les techniques permettant le développement de l’agriculture biologique.

en question l’indépendance de la recherche publique. En aucun cas des considérations ou intérêts économiques privés ne doivent interférer avec la qualité et la neutralité de cette dernière. Nous savons que les conflits d’intérêts existent déjà et que les grands groupes privés font pression pour influencer les études scientifiques, voire, dans certains cas, pour les produire eux mêmes, afin de brouiller au maximum le message vis à vis du grand public. Cet amendement n’est donc pas seulement sémantique : il reflète une réalité contre laquelle il faut lutter.

Ces collaborations devront être orientées vers les besoins en matière de transition agroécologique de notre agriculture. Nous y insistons fortement : si la recherche et l’innovation de notre pays ne se tournaient pas vers des modes de production plus durables et respectueux de l’environnement,

Il vise à préciser que les compétences à acquérir portent également sur les transitions agroécologiques et climatiques. Nous regrettons fortement que les rapporteurs aient supprimé cet objectif, qui nous paraît pourtant indispensable,

agricoles dans les domaines de l’agroécologie, de l’agriculture biologique ou encore de la transition climatique et environnementale, pour reprendre le dispositif de l’amendement du Gouvernement. Je rappelle que la rédaction actuelle vise notamment à accroître les connaissances des personnes formées dans le domaine de l’adaptation au changement climatique. La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception

l’effort de renforcement des connaissances devra également porter sur les domaines et techniques liés aux transitions climatiques et environnementales. De même, l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances

aux agriculteurs pour faire face au changement climatique est considérable et n’a rien à voir avec la révolution de la mécanisation agricole. Cela requiert Cela requiert une élévation du niveau de connaissances, de compétences et implique de savoir comment ils pourront exercer un métier que la transition climatique et environnementale va très profondément affecter et faire

amendement a pour objet d’indiquer, de façon générique, les principaux blocs de compétences que les actifs de l’agriculture et de l’agroalimentaire doivent développer grâce à la formation tout au long de la vie, pour être armés face aux enjeux de leur métier. enjeux de leur métier. Cet amendement est dicté par le souci de lisibilité de l’article programmatique. Nous préférons mentionner ces blocs de compétences à un seul endroit, qui concerne le niveau de formation.

le renouvellement des générations. Il est regrettable qu’il ne soit jamais mentionné dans le projet de loi. L’activité agricole est, par nature, cyclique, les productions étant organisées en fonction des saisons. pour répondre aux besoins lors des récoltes, tailles et traitements, les exploitants agricoles ont recours aux travailleurs saisonniers. Ces derniers font partie intégrante du modèle agricole. Afin de fidéliser cette main d’œuvre dans un secteur identifié parmi les secteurs en tension, nous souhaitons que les travailleurs saisonniers soient davantage incités à suivre des dispositifs de formation, d’autant qu’ils peuvent devenir de potentiels repreneurs d’exploitation.

: La parole est à M. Bernard Buis. Cet amendement vise à améliorer l’état de la recherche variétale consacrée aux légumineuses en France, qui constitue à ce jour le principal frein au développement de ces dernières. Aujourd’hui, la raison majeure pour laquelle de nombreux agriculteurs ne souhaitent pas se lancer dans la culture des légumineuses est le rendement peu élevé de cette

Les dernières lois de finances n’ont pas permis d’inverser la tendance. C’est pourquoi, avec cet amendement, et tout en reconnaissant le rôle de l’enseignement agricole privé dans la formation des actifs, nous portons une attention spécifique à l’enseignement agricole public, qui représente un véritable atout pour nos territoires et qui offre les meilleures garanties en termes d’accessibilité pour l’ensemble des élèves. Ce qu’il faut à notre pays pour répondre au grand défi du renouvellement des générations, c’est une formation publique gratuite pour toutes et tous,

Si nous voulons assurer le renouvellement des générations en agriculture et satisfaire nos besoins en termes de souveraineté, une place importante doit être accordée à cette question de la reconversion professionnelle.

La recherche publique a un rôle crucial à jouer dans le changement des pratiques agricoles. L’Inrae est un leader mondial de la recherche spécialisée en agriculture. Les travaux de l’organisation scientifique en faveur d’une transition vers des systèmes agricoles et alimentaires durables permettent de replacer l’agronomie au cœur du métier d’agriculteur. Pour ces raisons, il apparaît essentiel que l’Inrae participe pleinement à la rédaction de ce programme éducatif et contribue à assurer la promotion de nouveaux modèles de production fondés sur l’innovation et la durabilité. Quel

une sixième année d’approfondissement dans les territoires d’élevage, en particulier à Limoges, mais pas seulement, afin de favoriser l’ancrage territorial et le désir de s’installer sur des territoires qui ont besoin de vétérinaires supplémentaires. Il s’agit là d’une démarche originale, puisqu’elle

une région d’élevage. Certes, je sais que ce n’est pas le développement des formations vétérinaires qui contribuera à résoudre le problème, mais l’accompagnement des éleveurs me paraît d’autant plus nécessaire que nous assistons à une complexification des des prophylaxies. Autrement dit, il y a sûrement lieu de travailler à de meilleures relations entre les praticiens vétérinaires et les éleveurs. Pour ces

Sans biodiversité, pas d’agriculture : les enfants doivent être sensibilisés dès leur plus jeune âge au rôle essentiel des pollinisateurs, de la vie souterraine, des auxiliaires des cultures, des oiseaux spécialistes des milieux agricoles, prédateurs naturels de nombreux ravageurs. Quel

de troisième et de seconde sur les métiers du vivant. Il s’agit d’une bonne réponse, comme les travaux du Sénat l’ont montré à de nombreuses reprises. C’est en effet une sphère professionnelle qui demeure très mal connue de l’éducation nationale,

Nous avons en tête les difficultés importantes qu’ont rencontrées de nombreux jeunes de seconde en juin dernier ; le constat est similaire pour les élèves de troisième. La décision ministérielle n’avait été suivie d’aucune coopération entre les différents acteurs à même de garantir une mise en œuvre satisfaisante

que vous proposez, la promotion du programme national d’orientation et de découverte des métiers du vivant serait à destination de tous les élèves, autrement dit une cohorte de 800 000 personnes. Je vous laisse imaginer la campagne de communication qu’il faudrait lancer

des affaires économiques a souhaité utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir les métiers du vivant et les formations. Pourquoi pas ?

par la signature de conventions particulières. Il s’agit de promouvoir l’enseignement technique et supérieur agricole de façon à faciliter les relations avec l’éducation nationale et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment en matière d’orientation scolaire et étudiante. Quel

L’installation en apiculture subit un très fort ralentissement lié à des questions environnementales et sanitaires majeures entraînant des pertes importantes de colonies d’abeilles et à une concurrence déloyale sur le marché mondial du miel. Ce projet de loi doit être l’occasion de promouvoir et d’accompagner la formation professionnelle

J’ai eu l’occasion de m’exprimer hier sur le sujet, puisque d’autres amendements visaient à compléter des listes de métiers ou de secteurs d’activité par le mot « apiculture

en son âme et conscience cet amendement, ainsi nous formerons et nous sensibiliserons à l’agriculture, à l’élevage, à l’aquaculture, à la viticulture et…

440 collectivités proposent un PAT, dont l’objectif est de fédérer tous les acteurs concernés autour des enjeux liés à l’alimentation et donc à l’agriculture. Leur permettre de nouer des liens avec les acteurs de l’enseignement et de la formation est évidemment

à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires et au développement de la consommation de produits issus de circuits courts

de mobilisation des établissements d’enseignement technique agricole publics et privés liés à l’État par un contrat. Les auteurs de cet amendement estiment en effet que ce représentant ferait doublon avec celui qui est prévu à l’article 3. Nous serons donc très attentifs aux propos de Mme la ministre sur ce point précis afin de déterminer s’il y a vraiment lieu de supprimer ledit alinéa. Dans cette attente, nous proposons, par cet amendement, de le réintroduire dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale. Toutefois, par souci de transparence,

rétablir un alinéa supprimé en commission par MM. les rapporteurs. Il s’agit, plus précisément, de créer « un programme spécifique d’orientation et de découverte des métiers des professions de vétérinaire et d’assistant vétérinaire », à destination des apprenants. MM. les rapporteurs jugent nécessaire de rationaliser le nombre de plans

cet amendement, nous tentons d’apporter une réponse supplémentaire aux enjeux de renouvellement des générations d’actifs agricoles. Il s’agit, plus précisément, d’étendre le public concerné par une formation professionnelle aux métiers de l’agriculture et de promouvoir davantage les métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires.

le taux de récidive. Ainsi, nous demandons au Gouvernement un rapport évaluant les bénéfices et limites du développement de l’insertion sociale et professionnelle de personnes détenues en fin de peine une offre de formation dans les exploitations agricoles.

il est souhaitable que l’enseignement agricole promeuve les valeurs républicaines, qui sont le socle de notre communauté nationale et les conditions de sa cohésion. Aussi, cet amendement tend à préciser que l’enseignement agricole a pour mission de transmettre les valeurs de la République.

doivent maîtriser des compétences très spécifiques. Or la formation à ces métiers se heurte à plusieurs difficultés. Ainsi, le réseau de centres de formation, qui est en développement, peine à adapter ses programmes aux besoins réels du terrain. On déplore de ce fait un manque d’accès à la formation continue, en particulier pour les saisonniers. Notre amendement vise à mieux faire connaître ces enjeux et à inclure le pastoralisme dans les dispositifs d’information à destination des enseignants, afin que ces derniers puissent sensibiliser leurs élèves à ces métiers essentiels, mais souvent méconnus, dans les territoires.

Levier fondamental d’adaptation au changement climatique autant qu’aux aléas économiques, la diversification est pourtant peu mise en œuvre. Elle doit s’articuler autour de deux orientations. La première est la formation des agriculteurs dans les métiers de l’hydrologie, de l’agronomie, de l’apiculture, mais aussi de la conduite du changement nécessaire à l’agriculture de demain. est la restructuration des filières et l’adaptation du système économique, afin qu’il soit à même d’absorber les produits issus des nouvelles pratiques agricoles. si nous voulons donner une nouvelle orientation à notre système agricole, nous devons renforcer l’attractivité des métiers du vivant. Quel

En vertu du plan Enseigner à produire autrement, l’agroécologie est déjà intégrée aux référentiels de formation. Le manque constaté aujourd’hui sur le terrain concerne avant tout l’enseignement en agriculture biologique, qui constitue le modèle le plus abouti en matière d’agroécologie. L’agriculture biologique repose sur un cahier des charges et sur des référentiels de production clairement définis et exigeants. Inscrire dans la loi l’enseignement des modèles de production agroécologiques et en particulier de l’agriculture biologique est essentiel pour permettre aux élèves de l’enseignement agricole

et capacité de choix aux futurs exploitants. L’agriculture biologique et l’agriculture de conservation des sols sont considérées comme les modèles les plus aboutis en matière d’agroécologie. Leur promotion apparaît comme une perspective d’adaptation durable qu’il faut inscrire dans les orientations de l’enseignement et dans la formation professionnelle agricoles.

de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la nature et des territoires. Il s’agit d’y intégrer spécifiquement, aux côtés de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations, de la compétitivité de la diversité des systèmes de production, le développement de l’agriculture biologique. La France doit se donner réellement les moyens d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés dans ce domaine. L’enjeu de la formation initiale et continue à l’agriculture biologique, et de manière plus générale à la transition agroécologique, est fondamental si nous souhaitons réellement engager un changement de modèle. C’est en formant les futures générations à tous les types d’agriculture sans les opposer entre eux que nous pourrons relever l’ensemble des défis qui se présentent à nous. Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain étant particulièrement attachés au respect de notre objectif d’atteindre 21 % de la SAU en bio d’ici à 2030, ils préconisent d’intégrer spécifiquement l’enjeu du développement de l’agriculture biologique dans la loi.

et de la formation professionnelle publics. Notre groupe a défendu en séance publique le 15 février 2024 une proposition de loi visant à préserver les sols vivants, qui sont des milieux fragiles, mais ô combien essentiels à la vie

Cette réalité nous montre les limites du système actuel et de la manière dont la préservation des sols est prise en compte. Il est donc indispensable de mettre en œuvre de véritables politiques publiques, afin de préserver et restaurer les fonctions écologiques des sols, mais aussi reconnaître et défendre les services écosystémiques qu’ils rendent. La sensibilisation et le renforcement de la formation des nouvelles générations à cet enjeu spécifique apparaissent essentiels

ans après le lancement du premier plan Écophyto, qui visait déjà à une diminution de 50 % à l’horizon de dix ans, aucune baisse de l’usage des pesticides n’a pu en effet être observée. Dans le même temps, la santé des sols se dégrade et les pollutions de nos masses d’eau s’intensifient.

au sein des commissions professionnelles consultatives de

dispensent des formations contenant des modules d’enseignement spécifiques liés à la transition agroécologique et climatique, ainsi qu’à l’agriculture biologique. Cet amendement vise ainsi à prévoir la participation des représentants de la communauté éducative et de la société civile à l’élaboration des programmes et référentiels de formation dans les commissions professionnelles consultatives de l’agriculture.

des modules d’enseignement spécifiques et obligatoires liés à l’agriculture biologique. Ces dispositions permettront notamment de mettre en cohérence les missions de l’enseignement agricole avec les objectifs des plans gouvernementaux Enseigner à produire autrement,

nous ne fassions aucun effort pour assurer une offre de formation à la mesure de cet objectif. Les formations bio, qui exigent l’acquisition de compétences techniques et agronomiques bien spécifiques, ne représentent que 5 % de l’offre de formation actuelle dans l’enseignement agricole public. L’objectif des politiques publiques agricoles est d’encourager les pratiques agricoles les plus vertueuses pour assurer la transition agroécologique et l’installation d’une nouvelle génération d’exploitants au fait des problématiques environnementales et climatiques, au cœur des métiers du vivant.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à garantir un nombre minimum d’heures consacrées à l’agriculture biologique dans le parcours de toute personne formée dans l’enseignement agricole.

vise à supprimer une phrase redondante relative au partenariat entre les parties prenantes de l’enseignement agricole. Plusieurs dispositions allant dans ce sens existent déjà. Je pense à la mission d’animation de développement des territoires, quatrième mission de l’enseignement agricole, à la désignation d’un correspondant départemental de l’enseignement agricole, qui figure à l’alinéa 4 de l’article

à ajouter une septième mission tournée vers la transition agroécologique. Nous y sommes naturellement défavorables.

pour cette profession, qui est souvent insuffisamment développée chez les jeunes diplômés de l’enseignement agricole. Cette compétence est notamment cruciale pour sélectionner les végétaux les mieux adaptés à leur milieu et pour appliquer les techniques d’entretien les plus respectueuses de la biodiversité. Par souci de transparence, je précise que cet amendement reprend une demande de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep).

à M. le rapporteur. Cet amendement vise à conforter la vocation pédagogique des exploitations agricoles des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles

Cet amendement vise à mieux intégrer les établissements agricoles dans les projets alimentaires territoriaux (PAT). Ces derniers sont des initiatives locales qui rassemblent différents acteurs – agriculteurs, collectivités, associations, entreprises pour favoriser une alimentation locale, durable et de qualité. Ils permettent de renforcer le dialogue entre les agriculteurs et la société, de mettre en lien les producteurs et les consommateurs à l’échelle d’un territoire. À l’heure actuelle, les établissements agricoles sont seulement incités à participer à ces projets ; ce n’est pas suffisant. Nous proposons de renforcer leur rôle en les impliquant

de construire son parcours en fonction de son projet professionnel. En intégrant le bilinguisme dans la formation des jeunes, nous répondrions à plusieurs enjeux importants. Nous pourrions ainsi adapter l’enseignement agricole aux réalités et aux exigences professionnelles actuelles, dans un secteur où l’internationalisation et l’échange de savoir faire sont de plus en plus cruciaux. La maîtrise de plusieurs langues est un atout indispensable pour nos futurs professionnels, qu’ils travaillent à l’échelle européenne ou internationale. De plus, la formation des élèves serait enrichie. Ils se verraient offrir davantage de souplesse et de choix pour leur parcours, conformément à la philosophie de la réforme du lycée.

en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, d’apprentis, d’étudiants, de stagiaires et de personnels ». Michel Rocard a introduit très tôt, dans cette cinquième mission, une dimension internationale.

et nos cultures locales. La

au sein des parcours de formation agricole. Sensibiliser les futurs agriculteurs aux pratiques agroforestières permettrait de mieux faire comprendre les nombreux bénéfices des haies, sur les plans tant écologique qu’agronomique. ci jouent un rôle crucial dans la préservation de la biodiversité, la protection des sols contre l’érosion, la régulation des ressources en eau et la captation du carbone. Par ailleurs, elles contribuent à améliorer les rendements agricoles en favorisant les interactions positives entre les cultures et les écosystèmes naturels.

D’après la Fédération nationale de l’agriculture biologique (Fnab), si nous souhaitons atteindre notre objectif de 21 % de la SAU en bio, il faudrait créer près de 200 000 emplois. Par ailleurs, selon les régions, entre 30 % et 50 % des candidats

de l’enseignement agricole public, et ces formations sont inégalement réparties sur le territoire et au sein des cursus. L’objet du présent amendement est donc d’intégrer cette formation renforcée au sein des établissements, publics comme privés.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement a demandé que la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique soit reportée du mercredi 12 au jeudi 13 février, le matin, en premier point de l’ordre du jour. Il a également demandé l’inscription à l’ordre du jour du jeudi 13 février, en deuxième et troisième points, des lectures, sous réserve de leur dépôt, des conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet projet de loi d’urgence pour Mayotte et sur la proposition de loi portant diverses mesures visant à adapter le fonctionnement des instances de gouvernance des chambres d’agriculture et de la mutualité sociale agricole. Acte est donné de ces demandes. Pour chacun de ces textes, nous pourrions fixer le délai limite des inscriptions des orateurs des groupes le mercredi 12 février à quinze heures. Y a t il des observations ?… Il en est ainsi